filière a besoin d'une baisse urgente de charges. À La Réunion, par exemple, ce secteur va mal ; quelque 30 % des entreprises liquidées ou placées, chaque mois, en redressement judiciaire sont des entreprises du BTP.

favorable ; en effet, il assure une exonération complète jusqu'à 1,3 SMIC, puis dégressive jusqu'à 2,2 SMIC. Ce régime permet sans doute de couvrir une proportion importante de la rémunération des personnes employées dans le secteur des BTP. Le Gouvernement pourra peut-être apporter des précisions chiffrées sur l'évolution des cotisations et contributions sociales de ce secteur, dans les collectivités ultramarines concernées, mais, en l'état actuel de ses informations, la commission a émis un avis défavorable

Le barème de compétitivité renforcée a été mis en place, avec deux objectifs : favoriser les secteurs fragiles dans un contexte de concurrence internationale et contribuer au rattrapage en matière d'infrastructures de base, à la modernisation des entreprises et à la transition écologique. Ainsi, pour les secteurs éligibles à ce barème, les exonérations sont totales jusqu'à 1,7 SMIC, puis dégressives jusqu'à 2,7 SMIC. Les premières évaluations menées sur l'impact de la réforme pour les secteurs éligibles au barème de compétitivité renforcée ont montré que certains employeurs de ces secteurs ne bénéficiaient pas d'un niveau d'exonérations supérieur à celui de l'année précédente, et ce, alors que le Gouvernement s'était engagé à mettre en oeuvre cette réforme à périmètre constant.

Si ce dispositif représente un coût non négligeable de 36 millions d'euros, il reste insuffisant pour combler les pertes suscitées, estimées à 60 millions d'euros, dont 19 millions d'euros pour les seules entreprises guyanaises.

applicables aux entreprises intégrées dans le barème dit « de compétitivité renforcée ». Ainsi, le seuil de début de dégressivité linéaire serait porté de 1,7 SMIC à 2,2 SMIC et le point de sortie passerait de 2,7 SMIC à 3 SMIC.

la loi de financement de sécurité sociale pour 2019 a opéré un recentrage des exonérations sur les bas salaires, à un niveau proche du SMIC. Si les bas salaires correspondent bien à une part importante des rémunérations outre-mer, il convient de ne pas encourager une structuration de l'économie autour des métiers peu qualifiés, qui induirait une fuite des cerveaux. Les économies ultramarines souffrent d'un déficit d'encadrement et d'ingénierie, et il convient au contraire d'y attirer les professions qualifiées, en particulier dans les secteurs les plus exposés à la concurrence. Par surcroît, des simulations conduites depuis l'entrée en vigueur des règles actuellement applicables montrent que ces dernières ont entraîné une perte de compétitivité pour les entreprises des secteurs exposés, du fait de l'augmentation de leurs cotisations, mesurée par rapport au régime dont elles bénéficiaient antérieurement. Le dispositif contenu dans le présent de dégressivité et d'extinction de l'exonération des cotisations patronales.

Cela couvre probablement une très forte proportion des rémunérations des employés dans les secteurs concernés. La commission estime raisonnable d'en rester à cet équilibre plutôt que d'aller encore plus loin, jusqu'à 3 SMIC. Elle a donc émis un avis défavorable

porter le barème de 1,7 SMIC à 2 SMIC en matière de compétitivité renforcée. Cela faisait suite à un arbitrage du Président de la République, rendu à l'issue de discussions avec les élus d'outre-mer. C'est un effort significatif que le Gouvernement consent pour renforcer

les Ultramarins sont passés d'une suppression de 9 points de CICE à une baisse des charges salariales sur les cotisations maladie de 6 points ; il y avait donc déjà une perte de 3 points.

met déjà en difficulté les entreprises ultramarines. C'est la raison pour laquelle certaines d'entre elles, dans les secteurs très divers que l'on est en train d'évoquer, demandent à revoir ces seuils à la hausse.

En échange, on nous a promis le Graal : un régime reposant sur deux piliers, la compétitivité et la compétitivité renforcée.

insistons autant. Je comprends les réformes entreprises par le Gouvernement pour sortir de ces situations de difficultés chroniques et trouver d'autres solutions ; mais nous avons

aux entreprises bénéficiant du régime d'exonérations de cotisations et de contributions patronales, dit « régime de compétitivité renforcée », propre à certaines collectivités d'outre-mer,

de toutes les travées, de tenir compte de la réalité économique et sociale de ces territoires, donc d'actualiser le seuil de début de dégressivité linéaire des exonérations, de 1,7 à 2,2 SMIC, ainsi que le seuil de sortie, de 2,7 à 3 SMIC. En effet, sur les territoires d'outre-mer, les entreprises des secteurs de l'agroalimentaire, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la recherche et développement ou de l'environnement ont vu leurs charges globales augmenter du fait de la réforme, entraînant des des conséquences irréversibles en termes d'emplois, alors que ces territoires ont vraiment besoin d'embaucher. Ce sont justement les entreprises qui auraient la possibilité d'embaucher qui sont les plus touchées.

renforcée. Cet amendement vise à faire bénéficier du barème dit « de compétitivité renforcée » les associations ultramarines oeuvrant dans la lutte contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales. la lutte contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales. Cette lutte étant l'une des grandes causes du quinquennat, la marge de manoeuvre financière ainsi dégagée permettrait à ces associations de mener plus d'actions de prévention. La Guyane et La Réunion sont en effet respectivement sur les première et troisième marches du triste podium des départements où les violences conjugales sont les plus nombreuses. À La Réunion, par exemple, sept plaintes pour violences conjugales sont déposées chaque jour ; les forces de l'ordre sont intervenues 6 000 fois à domicile en 2018.

propre à certaines collectivités d'outre-mer concerne surtout le secteur concurrentiel. Je ne vois vraiment pas pourquoi ces associations seraient privilégiées par rapport à d'autres.

: La parole est à M. Olivier Cigolotti. Les associations de sécurité civile forment chaque année plus de 400 000 personnes aux gestes de premiers secours. Si, demain, ces associations doivent augmenter leurs capacités de formation, afin de remplir les objectifs ambitieux que notre pays s'est fixés, l'action des intervenants bénévoles ne suffira pas et devra être renforcée par l'emploi de formateurs salariés, ce qui représentera inévitablement un surcoût important. Cet amendement vise ainsi à exonérer de charges sociales les associations agréées qui recruteront des formateurs salariés.

les emplois salariés de formateur aux premiers secours, donc pour les associations agréées de sécurité civile. Mais enfin, on pourrait en dire autant pour beaucoup d'autres associations ! Où s'arrêtera-t-on ?

existe déjà d'autres dispositifs de réduction du coût du travail qui sont spécifiquement destinés à l'emploi des formateurs occasionnels ; ainsi, les cotisations de sécurité sociale peuvent être calculées sur une base forfaitaire lorsque la durée de travail n'excède pas trente jours par an

Afin de limiter son impact financier, cette mesure est limitée aux entreprises de moins de onze salariés. De par leur taille, ces entreprises ont moins que les autres la capacité de compenser la mise à disposition d'un de leur salarié par une modification de leur organisation. ce dispositif permettrait de valoriser les entreprises qui s'inscrivent dans une démarche citoyenne, en soutenant l'engagement, et de lever une partie du frein financier à l'embauche d'un sapeur-pompier volontaire.

En effet, l'essence même d'une rupture conventionnelle est de faciliter la gestion des suppressions d'emplois par les employeurs : elle leur permet de rompre les contrats de travail sans avoir à justifier d'un motif économique. Vous avez introduit dans la fonction publique cette logique désastreuse pour remplacer les agents fonctionnaires par des contractuels au statut précaire. Comment ne pas interpréter cette mesure autrement que comme une volonté d'économies ? Comment ne pas voir que vous torpillez ainsi le service public ? Fidèles à votre politique, que nous dénonçons depuis le début de l'examen de ce PLFSS, vous étendez au secteur public le dispositif d'exonération sociale des indemnités applicable aux ruptures conventionnelles des contrats de travail des salariés du secteur privé. Vous poursuivez ainsi sur votre lancée dévastatrice pour notre système de protection sociale, cet article prévoyant que l'État ne compensera pas les pertes de recettes pour la sécurité sociale. L'exception est bel et bien devenue le principe, comme l'ont souligné, avec diplomatie,

Pourquoi ne pas revenir, à l'inverse, sur l'exonération des cotisations sociales dues sur les indemnités versées à l'occasion des ruptures conventionnelles dans le secteur privé ? Vu le nombre de ruptures conventionnelles signées chaque année- 437 700 selon Pôle emploi en 2018 -majoritairement sur l'initiative des employeurs, les caisses de la sécurité sociale ne s'en porteraient que mieux Vous comprendrez, mes chers collègues, que nous ne saurions adhérer à un tel projet. Le fil rouge de ce PLFSS est bien de continuer à vider les caisses de la sécurité sociale tout en cassant les services publics. Compte tenu des débats que nous avons depuis hier, chacune et chacun prendra ses responsabilités en toute connaissance de cause.

par un autre mode de financement que celui des cotisations sociales, en l'occurrence l'instauration d'une microtaxe sur les paiements scripturaux. Ah non ! Mais si, monsieur le président de la commission ! On le

on va totalement fiscaliser les ressources de la sécurité sociale au détriment des cotisations. On va ainsi créer un régime d'irresponsabilité et développer un assistanat qui ne correspond plus du tout à la philosophie des ordonnances de 1945, même si celle-ci doit évoluer.

ne sont pas acceptables en l'état. Nous ferions bien mieux de réfléchir à des mesures structurelles pour réduire le déficit de la sécurité sociale- Dieu sait si les pistes sont nombreuses

de la sécurité sociale pour 2020, qui prévoit d'exclure l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) de l'assiette des contributions et cotisations sociales. L'ensemble des revenus et des gains, fussent-ils seulement ponctuels, honorifiques ou de remplacement, devrait être fiscalisé au titre de l'imposition des revenus sans dérogations ou niches injustifiées. L'élargissement de l'assiette imposable est le préalable à une simplification et à une baisse des taux de notre système de prélèvements. Par cohérence, nous proposerons également un amendement de suppression de l'article 2 du pour 2020, lequel prévoit d'exonérer d'impôt sur le revenu l'ISRC créée par l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l'amendement

où les syndicats sont moins présents et les salariés plus précaires et vulnérables. De plus, contrairement à ce que voudrait faire croire- entre autres -le Gouvernement, les ruptures conventionnelles ne constituent pas une aubaine de mobilité ou de reconversion pour le salarié. Au contraire, comme le montre une étude publiée par la Direction de la statistique en février 2019, plus de neuf salariés sur dix ayant quitté « à l'amiable » leur entreprise se retrouvent à la case chômage. Deuxièmement, ces exonérations de cotisations vont encore réduire les ressources de la sécurité sociale.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article 9.

Nous proposons, par cet amendement, de supprimer le dispositif d'exonération de cotisations sociales sur les indemnités versées à l'occasion des ruptures conventionnelles dans la fonction publique. Une nouvelle fois, vous prétendez lutter contre le déficit de la sécurité sociale, alors même

vouloir aligner le secteur public sur le secteur privé, mais vous omettez de dire que ce sont les caisses de sécurité sociale qui vont en pâtir. Il s'agit d'une perte de recettes très importante.

décisions de non-compensation prises par le Gouvernement dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale créent artificiellement un déficit des comptes sociaux et font de la sécurité sociale une variable d'ajustement du budget de l'État, ce qui en change la nature.

de la Suisse, et ce pour les revenus fonciers encaissés en France. Toutefois, les Français non-résidents établis dans un pays tiers ne bénéficient pas de cette exonération, qui constitue une inégalité de traitement fiscal et une discrimination devant l'impôt et décourage l'investissement immobilier en France de tous ces Français non-résidents établis dans des pays tiers.

les revenus immobiliers de source française de nos résidents affiliés au régime obligatoire de sécurité sociale d'un État tiers à l'Union européenne autre qu'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Aucune norme supra-législative ne s'oppose à ce que tous les non-résidents ne relevant pas d'un régime obligatoire de sécurité sociale français soient placés sur un pied d'égalité. Contrairement aux auteurs de l'amendement n° 435 rectifié , notre collègue propose de ne pas rendre cumulatifs les critères de résidence et d'affiliation à un régime obligatoire français. Il ne lui paraît pas opportun d'appliquer aux revenus du patrimoine et de placements perçus par les non-résidents les règles applicables aux revenus d'activité et de remplacement. Un tel dispositif aurait pour effet d'exonérer de CSG et de CRDS sur les revenus immobiliers tous les non-résidents, y compris ceux qui relèvent d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. Concrètement, cela reviendrait à exonérer les personnes ayant effectué toute leur carrière professionnelle en France et qui s'expatrient en Espagne ou au Maroc, au moment de leur retraite. La solution envisagée par notre collègue Cadic dans l'amendement n° 353 rectifié n'emporte pas non plus l'adhésion de Richard Yung. Cet amendement tend non seulement à exonérer de CSG et de CRDS les non-résidents à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français, mais aussi à remettre en cause l'application de la jurisprudence dite « de Ruyter » en assujettissant de nouveau à la CSG et à la CRDS les résidents relevant du régime obligatoire de sécurité sociale d'un pays de l'Espace économique européen

la Caisse de prévoyance sociale, et leur domicile fiscal n'est pas en France. Pour autant, ils ne sont pas exonérés de CRDS et se retrouvent soumis à une double imposition. Cette inégalité de traitement est d'autant plus importante que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019

alors qu'ils ne bénéficient d'aucune prestation sociale en France. Ceux qui résident dans l'Union européenne, en raison du refus du Gouvernement de supprimer ces prélèvements, ont saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Ils ont ainsi obtenu de ne plus avoir à s'acquitter des cotisations de exemptés. Les Français résidant hors de l'Union européenne, eux, se sont vu refuser cette exemption. Ils continuent donc d'être soumis à cette cotisation de 17,20 %, qui s'ajoute à la retenue à la source et qui conduit à des prélèvements totalement confiscatoires de 37,20 % à 47,20 sur leurs revenus français, dès le premier euro, ou sur leur retraite française, sans bénéficier d'aucune couverture sociale, retraite ou de chômage. Il s'agit d'une discrimination insupportable et d'une véritable injustice. Il me paraîtrait normal que le Sénat soutienne tous les Français, y compris ceux qui ne résident

a été indiqué l'année dernière lorsque le nouveau régime a été mis en place, le principe reste de considérer la CSG et la CRDS comme des impôts

sur les revenus du capital les personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale d'un autre pays de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse. Je tiens à le souligner comme vous, monsieur le rapporteur général, c'est le critère d'affiliation à un autre régime de sécurité sociale européen qui détermine l'assujettissement ou non à la CSG et à la CRDS, conformément à la jurisprudence. Le critère de résidence n'est pas pertinent pour motiver une exonération de CSG. Les revenus dont il s'agit sont des revenus de source française, qui doivent également contribuer au financement de notre système de protection sociale, en vertu du principe d'universalité de l'assiette de la CSG. Si ces amendements étaient étaient adoptés, cela conduirait à exonérer de CSG les revenus du capital de personnes résidant à l'étranger, même lorsqu'elles restent affiliées à la sécurité sociale en France, ainsi que les revenus de personnes qui résident en France et y acquittent leurs impôts, mais qui sont affiliées à une sécurité sociale d'un autre État.

Il ne s'agit pas de cotisation, mais d'imposition de toute nature et le paiement de ces deux contributions n'est pas synonyme d'accès à un droit. C'est simplement une participation de chacun de nos concitoyens sur leurs revenus, de manière à financer le système de protection sociale.

s'appliquer à une personne qui n'en bénéficie pas. À l'évidence, il y a une contradiction entre le droit européen et l'interprétation du Conseil constitutionnel. Tant que l'on veut rester

c'est contraire au droit européen. La CSG finance la protection sociale et, au titre du droit européen, on ne peut pas y être assujetti si l'on n'en bénéficie pas. C'est très clair

! C'est la raison pour laquelle il y aura des condamnations si vous ne changez pas d'avis.

la CSG est un impôt de toute nature. Il est dû sur l'ensemble des revenus de source française, que l'on soit affilié au non, bénéficiaire ou non d'un droit. La France s'est mise en conformité avec la jurisprudence de Ruyter. Nous avons fait notre travail, et nous en resterons là.

En effet, alors que la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement- les salaires et les pensions de retraite, par exemple -a été augmentée de 1,7 point en 2018, pour compenser la baisse des cotisations sociales chômage et maladie, la CSG sur les revenus du capital a été accrue de 1 point

créerait un rendement supplémentaire de 3 milliards d'euros au profit des caisses de la sécurité sociale, donc au profit de chacun, ce qui permettrait notamment de financer la revalorisation, à hauteur de l'inflation, de toutes les prestations sociales, comme les pensions de retraite

ne seront que trop faiblement réévaluées. Par ailleurs, la mesure d'urgence économique et sociale réduisant la hausse de la CSG pour certains retraités n'est pas suffisante. Il convient en effet de revenir à la situation antérieure au 1 janvier 2018 et de dispenser tous les titulaires de pensions de retraite de cette hausse de la CSG, sauf à maintenir une rupture d'égalité entre les retraités. Nous avons, mes chers collègues d'autres occasions de trouver des recettes supplémentaires, nous vous l'avons prouvé, pour compenser la baisse des cotisations de chômage et de maladie. N'aggravons pas plus la situation des personnes retraitées qui ont contribué solidairement durant toute leur vie active au financement de notre système de protection sociale. Quel

Le passage à 8,3 % du taux de CSG sur les pensions s'est fait dans le cadre d'une réforme plus générale incluant la disparition de nombreuses cotisations des actifs. où il semble difficile de réassujettir les actifs à ces cotisations, il ne me semble pas possible de revenir au taux de 6,6 % pour l'ensemble des retraités.

Le Gouvernement avait fixé un seuil de 2 000 euros mensuels au-dessous duquel les retraités ne sont pas assujettis au taux de CSG revalorisé. Par cet amendement, il s'agit de retenir un seuil représentant le coût moyen d'une maison de retraite médicalisée, ce qui permettrait de redonner du pouvoir d'achat aux retraités.

Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd'hui la pension minimum, dont le montant est de 902 euros nets par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu'il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres. Appliqué à ces revenus fonciers, un taux réduit de CSG permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, qui constituent un complément de retraite, et non pas un investissement à caractère patrimonial. Par ailleurs, le dispositif de cet amendement ne vise que les retraités agricoles. Quel

de plus ! La plupart d'entre eux, même s'ils ne se bercent plus d'illusions, ne peuvent pas attendre si longtemps. J'ose espérer que, si cette réforme des retraites continue à patiner comme elle le fait, nous pourrons au moins évoquer

Ponctionner davantage les revenus des retraités, c'est méconnaître le rôle charnière que jouent, notamment, les jeunes retraités dans notre société. Ils aident très souvent leurs enfants,

les terres arables, les prairies, les zones humides ou même les forêts, n'est pas particulièrement avantageuse. Pour les agriculteurs à la retraite qui ont travaillé toute leur vie sur ses terres, ce patrimoine foncier est un complément de revenu indispensable, d'autant que, nous le savons tous, leur retraite n'a toujours pas été revalorisée. Notre collègue Sylvie Vermeillet évoquait des retraites agricoles d'un montant de 902 euros nets par mois. C'est parfois bien moins, nous l'avions vu lors de l'examen de la proposition de loi du groupe CRCE, que nous soutenions à l'unanimité. Nous avions alors été empêchés par le Gouvernement d'aller plus loin. Pour ces retraités agricoles, il est nécessaire d'adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres. L'alignement des taux des prélèvements sociaux pour ces revenus fonciers sur ceux qui sont appliqués aux retraités permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, à savoir celle d'un complément de retraite et non d'un investissement à caractère patrimonial. Il me semble légitime que ces revenus fonciers bénéficient des mêmes taux réduits de CSG

au Sénat, que le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye est tout à fait convaincu de la nécessité de donner un véritable coup de pouce aux pensions et aux retraités agricoles.

sur les revenus du capital. Je confirme à M. le rapporteur général que, pour le Gouvernement, la question du niveau des pensions de retraite, notamment dans le secteur de l'agriculture, doit trouver sa réponse dans la réforme systémique des retraites qui sera présentée dans les prochains mois. Arrêtez ! Vous

Oui, nous exigeons une revalorisation des petites retraites. Oui, nous attendons une revalorisation des retraites agricoles, notamment des petites retraites agricoles, et la prise en compte des conjoints. En tout état

à ce qui a été adopté dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale. En effet, nous pensons qu'il n'y a aucune raison d'alléger davantage la contribution patronale, sauf à reconnaître la volonté du Gouvernement et de sa majorité de grever toujours plus le budget de la sécurité sociale. Le dispositif concerné, dont l'objectif affiché est de fidéliser davantage les salariés et mandataires sociaux d'une société, contourne, en réalité, la vraie question, qui est celle de l'amélioration des conditions salariales et des conditions de travail. Si une Si une entreprise souhaite vraiment garder ses salariés, elle devrait avant tout songer à augmenter les salaires- c'est d'ailleurs ce que nous n'avons de cesse de demander au Gouvernement au travers des amendements que nous défendons depuis tout à l'heure. Elle peut également mettre en place des dispositifs réellement incitatifs, comme prévoir une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée ou associer de manière plus effective les salariés à la vie économique de l'entreprise.

donnant un bel exemple d'instabilité fiscale. Par ailleurs, la loi de finances pour 2017 a profondément revu le régime fiscal et social applicable aux bénéficiaires du dispositif. Ainsi, l'assujettissement aux prélèvements fiscaux et sociaux applicables aux salaires a déjà réduit fortement l'attractivité de ce dernier. Pour ces raisons,

qu'il en soit, je le retirerai sans difficulté si on me le demande. Je voulais simplement attirer l'attention de notre Haute Assemblée sur le caractère nocif et contre-productif de la C3S. Le Conseil d'analyse économique (CAE) a relevé cet effet nocif en série sur toute la chaîne de production des entreprises françaises : à chaque élément de la chaîne de production, la C3S pénalise la compétitivité de nos entreprises.

En contrepartie de la suppression de la C3S et des hausses d'impôt sur les sociétés et de TVA qui en résulteraient, il serait opportun de réduire, voire de supprimer certains allégements de charges patronales, notamment sur les salaires supérieurs à 1,6 fois le SMIC, dont l'efficacité n'est pas démontrée, et, ainsi, de compenser la perte de recettes pour la sécurité sociale. Quel

telle que ceux qui n'ont pas de capital à la fin de leur carrière peuvent basculer dans la pauvreté, alors même qu'ils ont travaillé toute leur vie. Le montant moyen de la pension versée à un agriculteur retraité est, en effet, inférieur au seuil de pauvreté et au montant du minimum vieillesse, puisqu'il s'élève à 766

visait à reporter cette réforme à 2020. Il s'agit d'assurer de nouvelles ressources à destination de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de concrétiser l'engagement

Parce qu'il n'est pas pensable d'attendre 2025, nous vous proposons de modifier le système actuel, afin de garantir des pensions décentes aux retraités agricoles. Pour ce faire, monsieur le secrétaire d'État, madame la ministre, nous sollicitons l'extrême bienveillance du Gouvernement et l'appui de l'ensemble de nos collègues.

la question de la revalorisation des retraites agricoles, qui est un vrai sujet, auquel, une fois de plus, monsieur le secrétaire d'État, je souhaite que le Gouvernement apporte des réponses immédiates.

d'État, je suis sûr que vous vous mordrez les doigts

et d'impôt sur le revenu du dédommagement perçu par les aidants familiaux au titre de la prestation de compensation du handicap s'applique aux revenus perçus ou réalisés en 2019.

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) vient de publier son panorama bisannuel de la santé, qui regroupe les données les plus récentes de trente-six pays, dont la France, touchant à l'état sanitaire des populations.

Interdire ne sert à rien, donc la mesure envisagée est plutôt bonne. Cela ne va pas tout résoudre, mais cela peut limiter l'entrée dans l'alcoolisme de certains jeunes. Ils ont de petits budgets, donc augmenter le prix rend l'accès à ce genre de produits plus compliqué. L'enjeu est bien de repousser la première consommation des plus jeunes. Devenir alcoolique résulte de nombreux facteurs : tout d'abord, le contexte, le fait de vivre dans une famille ou un milieu où la consommation d'alcool est élevée ; la génétique peut également jouer un rôle

les premiers produits consommés sont déterminants dans le parcours de l'addiction : un alcool peu cher et facilement accessible rend la consommation plus facile. Le mode

un peu celui de l'alcool : on peut en boire de plus grosses quantités sans s'apercevoir que c'est fort. Enfin, un marketing agressif vise prioritairement les jeunes et les femmes, conditionnant des usages qui peuvent conduire à la dépendance. La parole

faire état de quelques données utiles pour essayer de travailler intelligemment, c'est-à-dire de concilier une filière économique avec les impératifs de santé publique. Dans notre pays, quelque 10 % de la population consomment 58 % du volume total d'alcool, et environ 20 % en consomment 80 %.

la référence au règlement européen du 10 juin 1991 renvoyant aux « vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits vitivinicoles Les apéritifs aromatisés à base de vin sont issus de savoir-faire régionaux. L'aromatisation des vins est une tradition qui remonte à l'Antiquité. Songeons aux vins d'orange, aux vins de pêche, aux vins de Noël, aux vins aux noix, aux châtaignes de l'Ardèche ou à la cannelle de l'Isère. Que de poésie les vins aromatisés sont strictement encadrés par le règlement européen et la loi du 26 février 2014, qui actualise les règles de définition, de description, de présentation, d'étiquetage et de protection des indications géographiques des produits vitivinicoles aromatisés.

de celui-ci en matière de prévention des consommations nocives d'alcool, en cohérence avec les deux priorités fixées par le Gouvernement : les femmes enceintes et les jeunes. Elle est également engagée auprès de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité dans une démarche de communication responsable.

et dont nous ne comprenons pas bien clairement les contours. Réaffirmons un modèle de consommation responsable conciliant art de vivre et préservation de la santé de nos concitoyens

sur les produits présentant un taux de sucre de plus de 35 grammes par litre et un degré d'alcool inférieur à 12 degrés, soit les deux tiers des produits encadrés par le règlement européen. Mes chers collègues, 3 000 euros par hectolitre d'alcool pur, c'est un niveau de taxation supérieur à celui de la vodka

de kir et d'autres recettes régionales fabriquées par des sociétés françaises. Il s'agit de vins aromatisés, non de premix. Je suis sûre, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, que le Gouvernement ne soutient pas cette initiative. Si c'était le cas,

semble se fonder à la fois sur une méconnaissance de la nature des produits concernés et sur une erreur d'appréciation des bénéfices espérés en termes de prévention de l'alcoolisme chez les jeunes. L'aromatisation des vins fait vivre une tradition qui remonte à des milliers d'années. Les vins produits, qui nécessitent la mise en oeuvre de plus de 20 000 hectares de vignes, font partie d'une catégorie viticole bien précise et définie de longue date par le règlement européen du 26 février 2014. Les apéritifs aromatisés à base de vin ne procèdent donc pas d'un processus de seconde main ; ils sont issus de recettes parfois ancestrales et d'un savoir-faire régional

par les plus de 35 ans et à 61 % par les plus de 50 ans. Par ailleurs, une taxe sur des produits moins alcoolisés risque de favoriser fortement un report de la consommation vers des produits plus alcoolisés,

Les premix sont les boissons les plus prisées des jeunes après la bière et les spiritueux. Et après la bière ! J'entends certains contester ce fait, mais j'aimerais qu'ils démontrent

les grandes marques de premix à base de vins le reconnaissent elles-mêmes. Enfin, toutes les appellations d'origine protégée et indications géographiques protégées sont hors du champ d'application de la mesure. Voilà, mes chers Le marché des vins aromatisés reste très limité. Et alors ? Ce sont surtout des majors qui seront concernées par cette taxe, dont les vins aromatisés ne représentent qu'un quantum marginal du chiffre d'affaires. L'objectif est d'arrêter le développement de nouveaux produits clairement dirigés vers les jeunes. En effet, les packagings de ces nouvelles boissons sont très colorés et imagés, rappelant les confiseries et les fruits pour s'acheter une innocence.

ne repose en réalité sur aucune justification en termes de santé publique. L'objectif est de taxer les boissons alcoolisées mélangées avec du sucre ou des boissons sucrées.

qu'est le bon vin. Ce n'est pas une éducation au bon goût, c'est un avilissement du palais que de faire boire ces produits à des jeunes et de les habituer à l'alcool avec ce type de boissons. La présente taxe tente de mettre fin à cette dérive, comme celle qui, il y a des années, a mis fin aux premix à base d'alcool fort et a permis d'arrêter leur consommation délétère pour la jeunesse

500 000 hectolitres de vin par an. Vous n'êtes pas sans savoir que le solde de la balance commerciale française des vins et spiritueux affiche pour 2018 un excédent de 13 milliards

d'être dit, il n'y a pas que les grands crus dans la production viticole. Le problème est bien de dissuader les jeunes

mais cette taxe est une mesure de prévention. Il ne faut pas confondre prévention et éducation à la santé. Taxer des alcools comme les premix est une façon de dissuader les jeunes

Le scrutin est ouvert.

Personne ne demande plus à voter ?

Le scrutin est clos. J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.